afin de nous permettre de nous rapprocher des objectifs d'énergie renouvelable fixés dans la directive européenne sur les énergies renouvelables. Les augmentations prévues à l'article 60, du pourcentage cible dans l'essence à 7,7 % en 2019 et à 7,8 % en 2020, en 2020, sont beaucoup trop faibles et ne correspondent pas aux besoins de notre pays, au vu de l'enjeu de décarbonation des transports et des capacités de production de bioéthanol excédentaires en France.

d'incorporation d'énergie renouvelable dans les essences à 8,3 % en 2019 et à 8,9 % en 2020. De plus, pour permettre aux distributeurs de carburants de procéder à cette augmentation, il tend à ne plus soumettre au plafond de 7 % le bioéthanol issu des résidus des industries sucrières et amidonnières. La trajectoire proposée est réalisable

Une telle mesure, je le rappelle, favoriserait la bioéconomie française, fondée sur des productions agricoles locales- je dis bien « locales » et non sur des importations -, dans une logique d'économie circulaire.

et permet que cette incorporation additionnelle puisse être réalisée, soit à partir de biocarburants de seconde génération, soit à partir de coproduits de l'extraction du sucre, en compte simple. Les coproduits issus de l'extraction du sucre sont, dans certaines circonstances, susceptibles d'être en concurrence alimentaire. Pour cette raison, seuls les coproduits obtenus à certains stades du processus pourront être pris en compte, dans la limite d'un plafond de 0,2 % en 2019 et de 0,3 % à compter de 2020, et en compte simple au contraire des biocarburants de seconde génération.

bioéthanol, pour ce qui concerne l'éthanol issu de résidus, du plafond de 7 % imposé aux biocarburants de première génération, afin d'atteindre des taux d'incorporation de 8,3 % en 2019 et de 8,9 % à partir de 2020.

Avec le système de « bilan massique » de la directive sur les énergies renouvelables, de l'ester méthylique de palme peut être commercialisé sous cette appellation. Par ailleurs, ces biocarburants issus des « effluents d'huileries de palme et rafle qui sont des produits d'importation bénéficiant du double comptage et donc d'une priorité d'incorporation dans les carburants, vont remplacer les esters méthyliques issus des filières françaises du colza et du tournesol. Dans la mesure où les externalités négatives des effluents d'huileries de palme et rafle sont équivalentes, voire pires que celles du tallol et brai de tallol, c'est-à-dire les acides gras,

rectifié. Cet amendement vise à ce que les biocarburants issus d'huiles usagées éventuellement importées- je dis bien « importées » -ne puissent pas se substituer aux biocarburants avancés français, tels que le bioéthanol issu de marcs de raisins et de lies de vin. Cet amendement a pour objet de permettre l'incorporation dans l'essence de ces biocarburants produits à partir de matières ligno-cellulosiques ou de marcs de raisins et de lies de vin, au-delà du plafond des biocarburants de 7 %.

Ce report est justifié par la nécessité de préserver les équilibres économiques entre les différentes filières françaises de biocarburants. Nous avons la chance d'avoir en France ces deux filières. Elles ne s'opposent pas, pas, elles ne sont pas en concurrence avec le domaine alimentaire. Ces deux filières doivent être développées, comme je l'ai dit précédemment, et bénéficier d'un fort taux d'augmentation.

rectifié et II-915 rectifié. Les effluents d'huile de palme, à ne pas confondre avec l'huile de palme elle-même, et les rafles permettent la production de biocarburants de seconde génération, dont l'impact environnemental est moindre que celui des biocarburants agricoles traditionnels. il n'y a pas de risque de déstabilisation des filières nationales par ces produits, notamment du fait des contraintes techniques et économiques particulières. Enfin, ces amendements nous paraissent un peu fragiles juridiquement.

le présent projet de loi limite déjà par rapport au droit actuel le recours aux huiles usagées en vue de limiter les fraudes. Nous considérons qu'une baisse additionnelle, motivée par un objectif de maintien de l'équilibre des filières, ne serait pas justifiée et caractériserait une rupture d'égalité non conforme à la Constitution.

La réforme de la fiscalité des biocarburants que nous portons vise à promouvoir les carburants de seconde génération qui n'entrent pas en concurrence avec de la consommation humaine- j'ai bien noté qu'il y avait un débat sur ce sujet.

demande le retrait

les analyses -, 0,5 % seulement de la déforestation mondiale serait due à l'huile de palme et son remplacement par d'autres cultures augmenterait significativement la surface terrestre totale utilisée pour la production d'huiles végétales. selon ce rapport, c'est en évitant davantage de déforestation grâce à l'huile de palme que l'on obtiendrait- de loin ! -les plus gros gains pour la biodiversité. Le rendement de l'huile de palme est en effet beaucoup plus élevé que celui des autres huiles végétales. La remplacer risquerait de nécessiter plus de terres et conduirait également à déplacer l'impact de ces productions vers d'autres écosystèmes, comme les forêts d'Amérique du Sud ou la savane africaine.

La culture de l'huile de palme est une cause majeure de déforestation en Asie du Sud-Est. Elle contribue ainsi de manière importante aux émissions de gaz à effet de serre, principale cause du réchauffement climatique. Le développement de cette culture a, par ailleurs, conduit à une perte massive de biodiversité, en raison de la destruction de milieux naturels à son profit. Les biocarburants à base d'huile de palme présentant un bilan carbone extrêmement négatif,

conçue pour recycler un certain nombre d'huiles : des huiles végétales certifiées durables, comme l'huile de colza ou l'huile de palme, des huiles alimentaires usagées, par exemple les huiles de friture, ou encore des résidus d'huiles utilisées en cosmétique et des graisses animales. l'objectif est d'atteindre un niveau d'incorporation d'énergies renouvelables dans les transports de 10 % en 2020 et de 14 % en 2030. Une somme de 275 millions d'euros a été investie dans ce projet et 1 000 emplois, dont 250 emplois directs,

dispositif extrêmement large, qui couvre l'intégralité de la filière de l'huile de palme, sans ménager de sort particulier à l'huile de palme issue d'une filière durable, c'est-à-dire garantissant la non-déforestation, la prise en compte des terres agricoles ainsi que la protection de l'environnement et des espèces animales.

Cette rédaction de l'article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d'emplois et qu'elle participe activement à l'indépendance énergétique de notre pays

Cette rédaction de l'article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d'emplois et qu'elle participe activement à l'indépendance énergétique et protéique de notre pays,

en demander le retrait. Quel est l'avis du Gouvernement ? Je rappelle que le Conseil constitutionnel, en matière de fiscalité comportementale, effectue un contrôle particulièrement strict du principe d'égalité devant les charges publiques et vérifie, en particulier, que les différences de traitement sont en adéquation avec la modification des comportements souhaités. Dès lors que le recours aux biocarburants de seconde génération et aux huiles usagées est davantage positif pour l'environnement que ne le sont les biocarburants agricoles traditionnels, limiter les premiers pour préserver les seconds nous paraît remettre en cause la robustesse juridique de cet impôt.

premier signataire, dont l'expertise est reconnue sur l'ensemble de nos travées. Nous vous proposons de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d'appliquer aux méthaniseurs non agricoles les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises déjà prévues pour la méthanisation agricole.

amendement vise à autoriser les collectivités qui le souhaitent à exonérer, sous certaines conditions, les services publics gestionnaires d'un réseau de chaleur biomasse de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, au même titre que le photovoltaïque et la méthanisation. de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet aux communes d'être compétentes en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid. Dans un contexte de difficultés d'investissement des collectivités territoriales, les dispositifs actuels de soutien ne permettent plus de créer ou de développer des réseaux vertueux. proposons-nous d'étendre, sous réserve que les collectivités territoriales le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du code général des impôts aux installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse. Les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à ces articles ne s'appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale mise en oeuvre par l'administration centrale exclut d'ailleurs expressément les réseaux de chaleur de ces exonérations, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées et ne s'exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. En outre, il s'agit d'une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants. Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées montrent que le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics. Notre amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière,

au-delà du simple soutien à la valorisation des déchets agricoles par méthanisation : il s'agirait d'une forme de subvention à des entreprises industrielles, parfois même à certains géants du secteur. Quant à

En application de l'article 1609 du code général des impôts, une taxe affectée est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échange de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers. Cette taxe affectée, qui correspond à 0,75 % du montant des salaires, est recouvrée au profit de l'Association nationale pour la formation automobile et participe au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle. Elle bénéficie aux entreprises relevant de la convention collective nationale des services de l'automobile

Or les entreprises de la distribution de pièces et d'équipements pour l'automobile sont susceptibles de relever d'une autre convention collective, notamment de celle des commerces de gros.

des dispositifs de formation

est l'avis du Gouvernement ? Cet amendement a pour objet de limiter le champ d'application de la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour la formation automobile aux entreprises relevant de la convention collective des services de l'automobile. Or le périmètre de la taxe comprend l'ensemble des entreprises ayant une activité de réparation, d'entretien ou de pose d'accessoires, notamment. Exclure du champ de l'impôt certaines de ces entreprises sur la base de leur appartenance ou non à une convention collective ne serait pas justifié.

Si les arguments tenant à la complexité du dispositif, aux modalités de perception et au très faible rendement de ladite redevance sont bien sûr recevables, l'absence d'évaluation d'une telle suppression sèche appelle à la prudence.

L'expérimentation issue de la loi Brottes vise à assurer à toutes les personnes physiques un accès à l'eau potable pour leurs besoins essentiels dans des conditions économiquement acceptables. Le nombre d'habitants dont la facture d'eau et d'assainissement dépasserait le seuil d'acceptabilité, soit 3 % du revenu, est estimé à 2 millions. Ce n'est pas tolérable, alors que le droit d'accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires fait partie des droits humains L'expérimentation de la tarification sociale de l'eau répond au besoin d'identifier et de mettre en oeuvre des solutions efficientes pour garantir la jouissance de ce droit. Concrètement, cette expérimentation permet aux collectivités territoriales volontaires d'inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus des foyers, de prévoir l'attribution d'une aide au paiement des factures ou encore d'une aide à l'accès à l'eau.

en métropole et neuf outre-mer. En avril 2017, soit un an avant l'échéance fixée par la loi Brottes, seulement la moitié des projets étaient mis en oeuvre. Ce décalage s'explique par le temps nécessaire à l'État pour mettre en place le cadre général. Mes chers collègues, il y a urgence, car une expérimentation

Le présent amendement vise à exonérer de la taxe sur les HFC prévue à l'article 60 du projet de loi de finances les pompes à chaleur destinées au chauffage central et à la production d'eau chaude sanitaire. En effet, ces pompes à chaleur utilisent des énergies renouvelables et constituent, de ce fait, une alternative énergétiquement performante aux solutions de chauffage conventionnelles. Elles s'avèrent indispensables à la réussite de la transition énergétique et à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone. En particulier, elles sont un des éléments clés pour atteindre l'objectif actuel du Gouvernement qui est d'éradiquer les chaudières au fioul à horizon de 2027. 2027. Les pompes à chaleur, handicapées par le supplément d'investissement qu'elles exigent par rapport aux chaudières conventionnelles, bénéficient pour cette raison du crédit d'impôt pour la transition énergétique.

j'ai le sentiment que vous ne comprenez pas ce que nous disons. J'en suis très triste, parce que les choses nous paraissent simples, peut-être parce que nous les vivons sur le terrain. Je voudrais vous rappeler un mot que j'aimerais que vous n'oubliiez pas : bouquet. L'énergie de demain,

transmettent " si elles sont connues de l'opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés " . » C'est vraiment un appel à la bonne foi : si je ne connais pas les coordonnées, je laisse passer ... « Le présent amendement prévoit

Une amende de 7 500 euros par manquement constaté, c'est-à-dire par logiciel non sécurisé, est prévue. Initialement, cette sanction relative au non-respect de cette obligation à l'attention des commerçants était fixée à 5 000 euros. Elle a été rehaussée pour rendre plus dissuasif son manquement. Or ce montant apparaît toujours excessif et disproportionné s'agissant d'une amende fiscale, pour les commerçants dont le chiffre d'affaires est limité. En outre, l'instruction fiscale est parue tardivement. De même, cette sanction va à l'encontre de la volonté du Gouvernement, qui souhaite passer d'une culture de contrôle à une culture de l'accompagnement et du conseil. Aussi, pour que la sanction soit plus en adéquation avec les capacités économiques des plus petites entreprises, il est proposé de ramener ce montant à 5 000 euros par manquement constaté, comme voulu initialement par le rédacteur.

Appliquée depuis 1948 aux exploitants de salles de cinéma dans l'Hexagone et depuis 2016 en outre-mer, cette taxe est collectée par le CNC et redistribuée, redistribuée, d'une part, aux exploitants pour accompagner la modernisation de leurs salles et, d'autre part, aux producteurs de films pour soutenir la production audiovisuelle.

le taux s'élève à 3 %. L'actuel article 62 prévoit de porter ce taux à 5 % en 2019 et de le geler à ce niveau.

le taux de 3 % permet aux exploitants d'atteindre l'équilibre aux Antilles-Guyane en conservant toutes les salles. Si la participation des exploitants ultramarins à l'effort national de soutien à la production et à la modernisation des salles est indispensable, elle doit se faire à un niveau permettant de garantir la survie de toutes les salles de cinéma, particulièrement des plus petites. C'est pourquoi cet amendement vise à fixer le niveau définitif le niveau définitif de la TSA à 3 % en outre-mer, et je ne doute pas qu'il recueillera l'unanimité.

Le code général de la propriété des personnes publiques indique, en son article L. 2125-1, que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance, mais les articles suivants la nature de cette redevance ni si celle-ci doit nécessairement être acquittée sous forme monétaire. Aussi, les personnes publiques gestionnaires de leur espace public peuvent-elles abandonner des recettes en numéraire en contrepartie de prestations offertes par le débiteur de la redevance ? Bien évidemment, ces prestations seraient telles que le prix unitaire de la contrepartie serait public de manière que tout un chacun puisse vérifier que la valeur marchande des prestations offertes est au moins égale au montant de la redevance due. due. Ce serait un moyen de modernisation publique et peut-être aussi une réponse à certaines préoccupations des collectivités : elles sont encadrées dans leurs dépenses sans, pour autant, être limitées dans leurs recettes. Tel est l'objet de cette question.

les prestataires visés par la décision d'arrêter les décaissements ou encaissements en numéraire dans les trésoreries publiques, publiques, ni comment ceux-ci seront dédommagés, ni comment la sécurité de leurs personnels et de leurs clients sera assurée. Bref, cet article est vraiment imprécis, trop imprécis pour être adopté, alors que 530 000 encaissements en numéraire ont été réalisés en 2017 pour permettre aux particuliers de payer leurs impôts et 500 000 pour leur permettre de payer leurs amendes. Au-delà du caractère imprécis et insuffisant de cet article, nous estimons qu'il en l'espèce d'un démantèlement de l'État dans l'une de ses missions régaliennes les plus fondamentales. En ce sens, cette disposition nous paraît extrêmement dangereuse au regard de notre vision du rôle de l'État, notamment en termes de présence dans les territoires. Bref, moins on en fait faire aux trésoreries, plus on les ferme facilement.

de 200 euros, par exemple, chez un buraliste ou dans un bureau de poste, mais les commerçants ne sont pas soumis au même niveau de secret professionnel que les agents des finances publiques. Le paiement se fera-t-il de manière

Ils pourront encaisser, et uniquement cela. À aucun moment, il n'est question de leur donner compétence ou même une quelconque délégation pour pour mettre en place un échéancier, pour discuter d'un éventuel allégement ou de la majoration d'une pénalité. Il s'agit simplement d'avoir des points de contact sur le territoire pour

extrêmement attentifs à la fois aux prérogatives de la puissance publique et à la confidentialité, tout en ayant la volonté d'avoir plus de points de contact sur le territoire afin de faciliter la vie des contribuables. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables aux amendements de suppression. En réponse à Mme Lavarde, je veux dire que de rares exceptions prévoient qu'un contribuable puisse s'acquitter de telle ou telle contribution ou de telle ou telle redevance par des prestations en nature. À ce stade, le Gouvernement n'est pas ouvert à un élargissement des exceptions prévues, pas plus qu'il n'est ouvert à un développement de ce mode de paiement.

prévoit la fusion des trois annexes générales du projet de loi de finances portant sur les dépenses et les ressources en faveur de la protection de l'environnement, du climat et de la transition écologique et énergétique en une seule annexe, qui annexe, qui s'intitulera. Il nous paraît important que cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises selon les secteurs d'activité. Pourquoi ? Parce qu'il est évident

d'une proposition qui ferait avancer notre droit positif dans un sens qui me semble extrêmement utile. Cet amendement vise à tirer les conséquences, en ce qui concerne le processus législatif, du principe général d'ouverture des données publiques posé par l'article 1 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. L'article 2 de cette loi a ajouté les « codes sources » à la liste des documents administratifs dont la liberté d'accès est garantie par les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les administrations sont donc tenues de publier en ligne ou de communiquer ces documents à toute personne qui en fait la demande. L'article 4 de cette même loi a, quant à lui, créé un principe de communication des algorithmes, lorsque ceux-ci ont participé au fondement d'une décision individuelle, ce qui s'applique naturellement aux impôts. À ce jour, seules des initiatives ponctuelles ont été prises, essentiellement à la suite de décisions juridictionnelles : par exemple, la publication du code source de la procédure d'admission post-bac par le ministère de l'éducation nationale en octobre 2016, ou encore la publication du code source de l'impôt sur le revenu par la DGFiP en mars 2016.

Aujourd'hui, nous ne le pouvons pas ! D'une certaine façon, le citoyen ordinaire a des droits qui lui sont accordés par la loi dont le parlementaire ne dispose pas pour légiférer. Vous nous enfermez ou, plus exactement, l'Assemblée nationale- puisque c'est elle qui a refusé cette avancée -nous enferme dans une législation à tâtons, pour ne pas dire « à l'aveugle », alors que nous voulons légiférer en toute connaissance de cause et sans avoir forcément à solliciter de façon itérative l'administration fiscale pour lui demander des simulations nous permettant d'apprécier les dispositifs fiscaux que l'on nous propose de voter ou que nous souhaiterions nous-mêmes infléchir. Une telle modernisation de la façon de travailler serait bonne pour le Parlement, et donc bonne pour le pays.

Quel est l'avis de la commission ?

aux centres d'hébergement de personnes ou de familles en difficulté, ainsi qu'aux établissements ou services médico-sociaux assurant l'accueil de personnes en situation de détresse et atteintes d'une pathologie lourde. Quel est l'avis de la commission ?

est déjà largement appliqué aux établissements médico-sociaux, notamment pour les personnes âgées ou handicapées, les structures d'hébergement d'urgence dans le cadre de la politique sociale. L'extension de ce taux réduit à des établissements n'ayant pas l'hébergement pour objet premier ne nous paraît ni justifiée ni étayée juridiquement. Il n'est pas envisagé de l'étendre à de nouvelles structures.

comme, par exemple, la légalité de son installation et le contrôle de sa qualification professionnelle. L'article 64 prévoit une baisse des tarifs et une dispense de paiement de ces redevances auprès des chambres de métiers pour les artisans qui choisissent une forme juridique sociétale et les artisans commerçants.

les chambres de métiers et de l'artisanat ont déjà tenu leurs assemblées générales et ont adopté leur budget pour 2019, en intégrant le montant des redevances en vigueur. Enfin, les dispositions de l'article 64 n'ont pas été anticipées

de l'artisanat oeuvrent au quotidien pour la simplification des formalités des porteurs de projets de création d'entreprise, et elles entendent bien poursuivre cette mission tant les besoins d'accompagnement sont importants. S'il était adopté définitivement, l'article 64 les priverait de ressources essentielles.

l'AAH atteint actuellement 860 euros mensuels pour une personne seule. Il est à noter que les personnes handicapées ont d'importantes difficultés d'insertion, puisque seuls 6 % des allocataires de cette prestation sortent des minima d'une fin d'année à la suivante. Ayant une vision bien précise des difficultés rencontrées au quotidien par ces allocataires, le Gouvernement a néanmoins fait tout le contraire de ce qui avait été promis baisse de 5 euros par mois de l'APL, augmentation de la CSG, de la CRDS, baisse du coefficient de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH, afin de l'aligner sur celui du RSA, suppression du complément de ressources servant à compenser la perte d'autonomie des plus fragiles, suppression de la prime d'activité pour les pensionnés d'invalidité, pour les pensionnés d'invalidité, suspension de l'application des normes d'accessibilité dans le bâti neuf prévues par la loi Handicap

il semblerait que vous ayez enfoncé le clou avec le décret n° 2018-767 et l'arrêté relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs,

pour les retraités et les handicapés, qui voient au fur et à mesure leur pouvoir d'achat diminuer comme peau de chagrin. C'est pourquoi il convient de supprimer cette mesure de revalorisation de l'AAH, fixée à 0,3 % en 2019 et en 2020.

Le code de la sécurité sociale prévoit que les prestations sociales doivent faire l'objet d'une revalorisation annuelle qui prend en compte le niveau de l'inflation. La présente revalorisation ne permet donc pas d'augmenter le pouvoir d'achat des allocataires, mais simplement d'éviter qu'il diminue du fait de l'inflation.

le Gouvernement qualifie de mesure d'augmentation maîtrisée des prestations sociales. Nous ne sommes pas dupes : désindexer les allocations de l'inflation équivaut mécaniquement à une baisse de leur montant, et non à leur augmentation maîtrisée.

Ce nombre nous paraît trop élevé au regard de l'effectif actuel de la profession et, plus encore, au regard de son effectif futur, amené à se réduire en raison des effets du relèvement des seuils de désignation de ces commissaires. Sans préempter le débat en cours au Parlement sur le projet de loi PACTE, cette réforme devrait affecter l'organisation territoriale des CRCC des opérations de regroupements. Le présent amendement vise à neutraliser l'impact fiscal de ces opérations. À droit constant, celles-ci pourraient effectivement conduire au paiement de droits parfois élevés, alors même que la vocation et l'objet des patrimoines ne changent pas. ne changent pas. Il s'agit donc d'exonérer de tous droits, taxes et contributions, y compris de la contribution de sécurité immobilière, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une CRCC

n° II-185 rectifié. Cet amendement tend à recentrer le champ d'application de la réduction de loyer de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l'APL. Les plafonds de ressources sont fixés, chaque année, par arrêté. Ils permettront de délimiter, parmi les ménages bénéficiaires de l'APL, ceux à qui s'appliquera la réduction de loyer de solidarité. Les cas de ménages ayant des APL inférieures au montant de leur RLS sont sources de surcoûts pour les organismes, au-delà de l'économie budgétaire attendue de 800 millions d'euros environ. Ils représentent également un surcoût en termes de gestion, celle-ci s'avérant très complexe pour les bailleurs, mais aussi pour les CAF et les CMSA. En jouant sur les plafonds de ressources, il sera possible pour le Gouvernement de réduire très fortement le nombre de ces cas.

et au terme de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, il est nécessaire de modifier l'article d'équilibre au regard des votes intervenus au Sénat sur cette seconde partie, les règles d'examen du projet de loi de finances nous interdisant, comme vous le savez, de revenir sur le vote de la première partie.

je ne suis pas sûr, mais c'est un avis personnel, que cela soit une réelle économie. Ces votes conduisent à améliorer le solde budgétaire de 57 milliards d'euros et à nous placer- fictivement, vous en conviendrez, puisque personne n'imagine que l'État puisse fonctionner sans les sept missions que j'ai évoquées